que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce texte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 chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs qui s'expriment à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents, réunie le 1 décembre dernier.

générale, la parole est à M. le ministre. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, lorsque je vous avais présenté, en octobre dernier seulement, le projet de loi qui est devenu la loi du 10 novembre 2021, j'avais appelé à un effort collectif de vigilance sanitaire- la situation était alors pourtant beaucoup plus favorable compte tenu des risques de reprise épidémique liés à la période hivernale et à l'apparition probable de nouveaux variants. Un peu moins de trois mois se sont écoulés et vous voici réunis aujourd'hui afin d'examiner un douzième projet de loi consacré à la lutte contre la pandémie de covid-19.

Cette situation, aussi vertigineuse qu'elle puisse être, exige que nous prenions nos responsabilités avec sang-froid afin de poursuivre la gestion d'une épidémie sans précédent, qui dure depuis bientôt deux ans. Les Français ont été courageux, tout le monde s'accorde à le dire. Ils ont fait face et je veux leur rendre hommage parce que les sacrifices qui leur sont demandés sont colossaux. Je comprends la fatigue, la lassitude, mais j'ai toujours dit que cette crise sanitaire serait une épreuve d'endurance. Le texte qui vous est soumis renforce plusieurs mesures existantes, lesquelles nous ont d'ores et déjà

Aujourd'hui, malgré la présence d'un variant extrêmement virulent, si nous pouvons envisager de vivre le plus normalement possible, sans empêcher ou fermer massivement les activités du quotidien, c'est parce que nous avons le vaccin.

pas le pas. Restent, enfin, ceux que nous aurons du mal à convaincre par des mesures pédagogiques et par des entretiens avec des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, ceux qui pensent encore qu'on leur veut du mal en leur proposant un vaccin qui protège. Une partie d'entre eux se laissera peut-être convaincre par la mise en place du passe vaccinal, pour beaucoup, le registre rationnel a été mobilisé en vain. Toutefois, nous ne devons pas relâcher nos efforts. À court terme, de nouvelles mesures de freinage ont été décidées. Je pense notamment au nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine lorsque cela est possible, au port du masque à l'intérieur dès l'âge de 6 ans ou encore à la mise en place de jauges pour les spectacles culturels et les événements sportifs. Nous avons également décidé d'adapter les règles en matière d'isolement et de quarantaine, afin de tenir compte de la diffusion extrêmement rapide du variant omicron des données virologiques disponibles, mais également de maintenir la vie socioéconomique du pays et le fonctionnement des services publics. Sur le fondement d'un avis rendu par le Haut Conseil de santé publique le 31 décembre 2021, ces règles ont été harmonisées et simplifiées depuis lundi dernier. Enfin, et c'est précisément l'objet du présent projet de loi, nous souhaitons renforcer plusieurs outils de gestion de la crise sanitaire déjà prévus par la loi. Nous proposons ainsi un approfondissement des mesures de protection et la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal,

Après la promulgation de la loi, il sera donc nécessaire de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux débits de boissons, aux foires, aux séminaires, aux salons professionnels et aux transports interrégionaux.

Par ailleurs, le projet de loi renforce encore les mesures permettant de lutter contre la fraude. Nous savons combien la pratique des faux passes peut être dangereuse pour les personnes qui s'y adonnent. Toute personne habilitée à demander la présentation d'un passe pourra ainsi exiger également celle d'un document permettant de vérifier

Nous proposons également, et c'est important, que les services préfectoraux puissent connaître des données strictement nécessaires à leur mission de contrôle des mesures de quarantaine et d'isolement, afin de vérifier que chaque personne concernée a bien réalisé le test négatif conditionnant la levée

de renforcer l'intervention du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un régime de contention et d'isolement en psychiatrie. Le texte a été modifié par l'Assemblée nationale sur plusieurs points en matière de police sanitaire, afin de s'assurer du respect par les employeurs de leurs obligations de prévention, notamment en matière de télétravail ; pour adapter l'application du passe vaccinal aux mineurs ou encore pour faciliter l'engagement dans un parcours vaccinal des personnes ayant commis une fraude au passe sanitaire. loi a également été complété par plusieurs mesures visant à soutenir le système de santé, telles que la prolongation de la garantie de financement des établissements de santé et du dispositif d'indemnisation de la perte d'activité des médecins ; des adaptations des règles de cumul emploi-retraite pour les professionnels de santé ; la prolongation de la prise en charge à 100 % des actes de téléconsultation. Enfin, le texte qui vous est soumis réactive des mesures adoptées lors de phases précédentes de la crise sanitaire, qu'il s'agisse des règles de réunion des assemblées générales de copropriétaires, de la constitution des jurys d'assises ou encore de l'organisation des concours de la fonction publique. Le projet de loi a été significativement modifié sur l'initiative de votre commission des lois et de votre commission des affaires sociales. Parmi les principales modifications adoptées en commission, je relève en particulier que vous avez souhaité définir des seuils de déclenchement du passe vaccinal à l'échelon national ou, à défaut, à l'échelon local, en inscrivant dans la loi un nombre d'hospitalisations cible. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Vous avez également proposé d'exclure l'application du passe vaccinal aux mineurs, alors que l'Assemblée nationale avait souhaité en exempter les seuls 12-15 ans pour toutes les activités extra et périscolaires, de nature culturelle ou sportive par exemple. également souhaité exclure la possibilité d'appliquer le passe vaccinal ou le passe sanitaire aux centres commerciaux et aux grands magasins. Vous avez supprimé le dispositif inséré à l'Assemblée nationale, sur l'initiative du Gouvernement, visant à faciliter l'engagement dans un parcours vaccinal des personnes ayant commis une fraude au passe. C'est ce que l'on a appelé le droit au remords ou à la repentance, peu importe la terminologie. Vous avez écarté le dispositif de sanction adopté par les députés pour assurer le respect par les employeurs récalcitrants de leurs obligations de prévention en matière de santé et restreint la prise en charge à 100 % de la téléconsultation aux actes s'inscrivant dans un parcours de soins coordonnés. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces modifications lors de la discussion des articles. Les amendements présentés par le Gouvernement n'épuisent pas l'ensemble des sujets de discussion, mais nous avons souhaité nous concentrer sur les points les plus saillants à ce stade. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, le présent projet de loi ne bouleverse pas l'économie générale de la gestion de l'épidémie, mais il vient renforcer et enrichir les outils mobilisés pour maîtriser au mieux l'évolution de la situation sanitaire. Il demeure tout entier guidé par la recherche de cet équilibre difficile, avec le souci premier de protéger les Français,

À ceux qui sont certains d'avoir toujours raison, dans leurs raisons d'ailleurs successives, j'opposerai simplement mes propres doutes et les quelques convictions qui ont pu s'en détacher.

Mais je ne prétends pas exercer la police du langage ! La vitesse de propagation du virus est sans précédent. Paradoxalement, ce texte n'a pourtant pas pour objet de répondre à l'urgence sanitaire. Pour la quasi-totalité des Français, le passe sanitaire est déjà un passe vaccinal. nous disposons d'un arsenal législatif considérable, que le Gouvernement ne souhaite mobiliser qu'avec parcimonie. il s'est hâté avec lenteur depuis l'annonce faite par le Premier ministre, le 17 décembre dernier. Quand il avait fallu mettre fin à la crise des gilets jaunes en décembre 2018,

Depuis lors, le Sénat a constamment assumé ses responsabilités et s'est engagé dans la lutte contre l'épidémie en conjuguant exigence sanitaire, respect des libertés et contrôle parlementaire. Il a toujours accordé aux autorités sanitaires les pouvoirs nécessaires en posant ses propres conditions. C'est dire combien serait inacceptable toute mise en cause de notre esprit de responsabilité dans un contexte d'instrumentalisation politique de la lutte contre le covid par l'exécutif. Alors que nous sommes confrontés à 100

entrera en vigueur à partir de la mi-janvier, mais ne produira ses premiers effets qu'à partir de la fin du mois de février- il faudra du temps pour que les nouveaux convertis à la vaccination soient pleinement protégés -n'est en aucun cas à la hauteur du problème.

Il est vrai que, sans que l'on puisse encore en déterminer la mesure exacte, le variant omicron, qui évince désormais le variant delta, semble beaucoup moins offensif et ouvre l'espoir d'une sortie du tunnel épidémique. Je veux le croire ! Mais ici et maintenant, nous sommes confrontés à une urgence sanitaire à laquelle le passe vaccinal, aussi utile qu'il puisse être, ne répond pas. Le désordre à l'école, dans le travail et, surtout, à l'hôpital, auquel le Gouvernement n'a pas préparé le pays, ne sera pas réparé par des imprécations contre les non-vaccinés, qu'il faut convaincre au lieu de les montrer du doigt, au risque de les braquer Je suis fermement partisan de la vaccination, et ce depuis le début ! Elle a déjà sauvé de nombreuses vies humaines et elle en sauve encore tous les jours. Ses effets indésirables doivent être rapportés au risque épidémique auquel nous sommes confrontés, que le vaccin réduit sans pouvoir l'éliminer. Il y a un large consensus médical en faveur du vaccin. S'il y a des voix scientifiques discordantes, auxquelles il convient, bien sûr, de prêter attention, il n'y a pas de choix plus raisonnable que de s'appuyer avec humilité sur ce consensus, d'autant que les résultats positifs du vaccin pour la santé publique sont tangibles : il atténue fortement le risque d'être malade ou de développer une forme grave de la maladie. Ce sont des faits L'un des enjeux essentiels est donc bien aujourd'hui encore de convaincre les hésitants de changer d'idée sur la vaccination, d'abord pour eux-mêmes et pour leur famille, ensuite pour l'ensemble de la collectivité nationale. Mais comment faire ? Pouvons-nous imaginer réussir à convaincre ceux de nos compatriotes qui craignent le vaccin plus que le covid en les outrageant ? Ou même simplement en essayant de les circonvenir : Vaccinez-vous et vous pourrez aller au restaurant et au cinéma ! » Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais cela révèle une piètre opinion des Français que de leur mettre en main un tel marché. On ne peut à la fois faire appel à la responsabilité de chacun de nos concitoyens et les traiter de manière aussi infantilisante en situant l'ordre de leurs priorités de manière aussi dégradante. Beaucoup de nos compatriotes qui refusent le vaccin le font par conviction. Nous sommes en désaccord avec eux, sans doute, car ils se mettent en danger et leur imprudence aggrave les tensions sur notre système de soins fragilisé, mais comment faire évoluer leur conviction sans leur montrer d'abord un peu de respect ? Il n'est pas juste de les accuser d'être à l'origine de la flambée de l'épidémie, puisque les trois quarts des personnes actuellement contaminées sont vaccinées. On ne peut davantage leur reprocher de saturer l'hôpital, car les malades du covid hospitalisés en soins critiques sont pour près de la moitié des personnes vaccinées. Si l'hôpital est aujourd'hui sous tension, c'est dû à la fatigue collective d'une institution éprouvée par le covid ; c'est lié aussi aux contaminations au sein même des équipes de soins, mais ce n'est pas sans rapport non plus avec une politique hospitalière qui n'a commencé à s'intéresser à l'usure de notre système de soins qu'avec la crise sanitaire. De ce point de vue, les non-vaccinés ont bon dos En l'absence d'obligation vaccinale, les personnes non vaccinées sont donc dans leur droit, même si leur comportement soulève un réel problème de santé publique. Par conséquent, le seul argument médical possible en faveur du passe vaccinal, c'est l'argument de la protection et non celui de la punition. Nos compatriotes non vaccinés sont plus exposés que les autres à une forme grave de covid, surtout quand ils appartiennent à des catégories médicalement vulnérables. Ils ont donc un intérêt majeur

éviter de fréquenter les lieux qui les exposent le plus aux contaminations, à commencer par ceux où l'on mange et où l'on boit, parce qu'il n'est pas possible d'y porter un masque comme à cette tribune.

nous avons posé nos conditions et fait en sorte que l'exigence de contrôle de la représentation nationale soit respectée. Et nous avons refusé les chèques en blanc en imposant le retour devant le Parlement si les paramètres du passe sanitaire devaient évoluer. Nous y voilà de nouveau ! Ce débat législatif, que vous avez à toute force voulu éviter en octobre, lorsque nous avions fixé l'échéance de février, vous avez décidé de l'ouvrir en janvier Sans enthousiasme, je vais donc proposer au Sénat d'admettre ce durcissement du passe pour les motifs de protection sanitaire que j'ai énoncés, mais en assortissant notre accord de quatre conditions destinées à préserver les libertés et la responsabilité de chacun. Le maintien de ce passe ne sera pas laissé à la discrétion du Gouvernement actuel et de ceux qui le suivront jusqu'au 31 juillet, puisque le passe s'éteindra de lui-même progressivement au fur et à mesure que les critères que nous aurons posés seront réunis. Les entreprises accueillant du public ne seront pas contraintes d'effectuer des vérifications d'identité, mais seront en revanche protégées par la loi quand elles demanderont un document avec photographie pour vérifier qu'il correspond bien au passe. L'inspecteur du travail ne pourra substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la nature des postes « télétravaillables » ni infliger à l'entreprise de sanction pénale en fonction de cette appréciation. Les règles applicables aux mineurs de plus de 12 ans pour leurs sorties scolaires et extrascolaires seront simplifiées et unifiées. Pas de passe vaccinal en dessous de 18 ans Si ces conditions sont respectées, je vous demanderai, mes chers collègues, d'approuver les propositions de vos commissions. Nous adresserons aussi une double mise en garde au Gouvernement face à la déferlante omicron, il doit sortir d'une posture attentiste susceptible d'amplifier la crise et de désorganiser la société, l'école, l'hôpital et l'économie ; face à l'émotion causée par les propos blessants tenus par le Président de la République la semaine dernière, il doit réparer au plus vite les torts faits à la cause de la vaccination en renouant le fil du dialogue avec nos concitoyens non vaccinés. Dans ce domaine comme dans d'autres, il vaut mieux convaincre que stigmatiser ! C'est vrai ! Le Président de la République le sait d'ailleurs par expérience,

si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun ». On ne saurait mieux dire

les effets du variant delta et, depuis décembre, de la rapide propagation du variant omicron, conduisent notre pays à affronter une double vague épidémique. Face à celle-ci, et alors que la vaccination est aujourd'hui notre principal et plus efficace outil de lutte contre le virus, le Gouvernement nous invite à transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. L'objectif affiché est double : restreindre l'accès des non-vaccinés aux lieux identifiés comme étant propices à une contamination et les inciter par là même fortement à se faire vacciner. Il s'agit donc d'abord de protéger les non-vaccinés eux-mêmes, mais aussi de répondre à l'impératif fondamental qu'est la préservation de la santé des Français dans leur ensemble. Alors que notre système de soins est sous tension et que nos soignants sont épuisés, garantir la santé de nos concitoyens, c'est aussi prévenir des hospitalisations évitables grâce à la vaccination. aussi réduire les déprogrammations, la saturation de nos hôpitaux et, partant, limiter les pertes de chance. Si nous regrettons que le Gouvernement n'assume pas clairement une obligation vaccinale de fait, notre commission a choisi de soutenir l'adoption de ce nouvel outil. Parmi les articles dont la commission des affaires sociales s'est vu déléguer au fond l'examen, quatre prolongent des dispositifs dans le champ de la santé : l'article 1 prolonge la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des téléconsultations l'article 1 prolonge le dispositif d'aide aux médecins libéraux des établissements de santé ; l'article 1 ouvre la possibilité d'une nouvelle garantie de financement des établissements de santé pour le premier semestre 2022 l'article 1 étend une nouvelle fois la dérogation aux règles de cumul emploi-retraite pour les soignants. Notre commission des affaires sociales s'est montrée réservée sur les nouvelles dérogations proposées à la hâte dix jours après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, aurait légitimement pu les porter. Aussi, même si elle a validé l'essentiel de ces dispositions, elle a souhaité encadrer la nouvelle exonération du ticket modérateur, alors que le retour au droit commun doit pouvoir se faire pour les téléconsultations.

applicable aux employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention des risques d'exposition de leurs salariés à la covid-19, le recours au télétravail étant visé par le Gouvernement. Les employeurs, qui sont déjà soumis à l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de leurs salariés sous peine de sanctions pénales, se sont très largement mobilisés depuis le début de la crise sanitaire. La commission a rejeté cette nouvelle logique coercitive, qui n'apparaît ni utile ni souhaitable, et qui donnerait une trop large marge de manoeuvre à l'inspection du travail. Par ailleurs, l'article 1 prévoit un nouveau report des visites médicales qui doivent être assurées par les services de santé au travail dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs. L'accumulation des reports pouvant être préjudiciable, la commission a limité la portée de cette disposition aux visites et examens qui n'ont pas encore été reportés en application de précédentes mesures. En outre, afin de prévenir un risque d'engorgement des services de santé au travail à l'issue de la crise, nous avons renvoyé à 2023 l'entrée en vigueur de la nouvelle visite médicale de mi-carrière prévue par la loi du 2 août J'en viens enfin à l'article 3, relatif aux mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, qui vient pallier une triple censure constitutionnelle.

peut ordonner la mainlevée de la mesure ou autoriser son maintien. La commission a adopté cet article, mais a souhaité notamment préserver la liste actuelle des personnes informées quand de telles mesures

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Le Sénat que j'aime, c'est le Sénat qui a interrompu le funeste projet de déchéance de nationalité. Jalouse de son pouvoir législatif, la Haute Assemblée a toujours son histoire, au rendez-vous de la préservation des libertés publiques, y compris quand elle a dû brider l'exécutif et ses excès. Aujourd'hui, nous en sommes au douzième texte législatif en La caisse à outils n'est jamais assez complète ; à chaque fois, le Gouvernement vient demander au Parlement de la compléter. Ce faisant, nous avons pris le chemin sans retour de la limitation des libertés publiques ; nous devons nous poser maintenant la question de la marche arrière. Je m'y oppose, tout d'abord, en raison du passe vaccinal. Le variant omicron déferle sur la France et les personnes testées positives se comptent par centaines de milliers chaque jour, y compris, massivement, parmi les vaccinés - je sais de quoi je parle de s'interroger sur l'utilité des mesures privatives de liberté actuellement applicables dans notre pays. Pour cela, il nous faudrait des éléments objectifs et chiffrés, dont nous ne disposons pas, monsieur le ministre ! Je m'y oppose, ensuite, en raison des contrôles d'identité

Quel effondrement de la pensée et du débat politiques nous a conduits là ? Les résignés disent : « On n'a pas le choix ! » ; les penseurs ne voient pas le problème ; quant aux visionnaires, ils affirment que c'est non pas la loi qui limite les libertés, mais le virus Je m'interroge : où est la gauche des droits de l'homme ? Où est la droite des libertés ? Où sont les syndicalistes, les universitaires, les intellectuels ? Ils sont si rares, ceux qui rappellent le prix de la liberté Mes chers collègues, je vous propose donc de dire un non ferme et définitif à cette très mauvaise idée du passe vaccinal, qui nous conduit tout droit au contrôle social généralisé. Pour conclure mon propos, je citerai Tocqueville, monsieur le rapporteur. Cet État se veut si bienveillant envers ses citoyens qu'il entend se substituer à eux dans l'organisation de leur propre vie. Ira-t-il jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d'eux-mêmes ? Le plus grand soin d'un bon gouvernement devrait être d'habituer peu à peu les peuples à se passer de lui.

interdit par principe à la République, tellement attachée qu'elle est à l'État de droit fondé sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de restreindre ou de limiter temporairement des libertés pour faire face à une crise majeure ?

collègue, dans notre pays, patrie des droits de l'homme, toutes les libertés sont sacrées, mais aucune liberté n'est un absolu. absolu. Le fondement de la liberté dans notre pays, l'article IV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le dit bien : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

l'éradication de l'épidémie de covid-19. C'est pourquoi, mon cher collègue, quoique je vous aie écouté, comme toujours, avec beaucoup d'intérêt et d'attention, je ne peux pas partager le point de vue philosophique en défense de cette motion. Je dois vous dire que je préfère de beaucoup que notre assemblée, plutôt que de refuser le débat,

a obtenu que nos débats se déroulent dans de bonnes conditions, dans une temporalité mieux à même de faire émerger des positions argumentées et des contre-propositions réalistes. Oui, ce texte est dangereux, nous vous rejoignons, mon cher collègue, sur bien des points, mais notre opposition nous engage à en discuter. Il est essentiel que le Gouvernement écoute nos positions et nos propositions. Aussi, bien que nous comprenions les arguments en faveur de cette motion, nous estimons néanmoins que la tenue d'un débat est essentielle, nécessaire et plus que justifiée par l'ampleur des conséquences de cet état d'urgence sans fin sur notre pays.

saurait être franchie : celle des injures et, pire encore, des menaces, dont les auteurs doivent être rappelés au sens commun et, si nécessaire, à la loi. la loi. Notre impératif central, en tant que législateur, est d'écouter la science. Tous les cercles et les institutions légitimes, offrant les garanties de rigueur et de probité dans l'analyse de cette maladie, nous le disent : hormis certains cas de contre-indication à la fois rares et bien délimités, il est confirmé

les constatations de la Société française d'anesthésie et de réanimation font quant à elles apparaître un tout autre chiffre : environ 5

! Les risques induits par la fraude doivent donc être pris au sérieux. C'est pourquoi la vérification de la conformité de l'identité

Le risque d'être pris en faute réduira significativement le recours à ces faux passes, qui sont un véritable danger. Il nous semble donc qu'il convient de maintenir cette disposition prévue dans le texte Nous souhaitons aussi maintenir la faculté pour l'inspection du travail de prononcer des amendes administratives

Cette crise, encore en cours d'accentuation pour une période que j'espère limitée, met une fois de plus en lumière le courage des soignants et des autres professionnels des services au public : enseignants, personnels de sécurité, travailleurs de l'espace public, et j'en oublie. Ils sont un rappel vivant à notre obligation d'être vigilants et efficaces dans notre mission de législateur.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, contrairement à ce que prétendent depuis des mois les trafiquants de, les résistants des boulevards, les de la chanson française et les Sakharov de la dictature sanitaire, nous avons aujourd'hui trois certitudes premièrement, le vaccin empêche l'immense majorité des formes graves ; deuxièmement, la probabilité d'un séjour en réanimation est dix fois supérieure chez les non-vaccinés ; troisièmement, les services d'urgence sont remplis par la petite minorité qui refuse la vaccination. La conclusion est d'une simplicité biblique : il faut vacciner il faut vacciner le plus de monde possible, le plus vite possible. Cela, 92 % des Français l'ont compris, mais pas les antivax. Depuis un an, ils nous tannent avec leur « convaincre plutôt que contraindre » ; ils nous disent de faire de la pédagogie et de ne pas stigmatiser, eux qui stigmatisent tous les autres. Il faudra bientôt vacciner en cachette et raser les murs pour ne pas les déranger. Eh bien, nous n'allons pas raser les murs, nous allons répondre ! Nous répondrons aux politiciens aux abois qui essaient de se refaire la cerise, aux philosophes de comptoir qui confondent liberté et irresponsabilité, aux agités du télébocal qui crient à la démocratie bafouée ! Nous répondrons aux Philippot, Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan ou Mélenchon, ce pacte germano-soviétique de la désinformation ! Ils ont été successivement pour la chloroquine, contre le vaccin, contre le passe sanitaire et maintenant contre le passe vaccinal, avec une infaillibilité absolue dans l'aveuglement. Ces amoureux des dictatures, il faut quand même qu'ils soient gonflés pour accuser le Gouvernement et le Parlement de prendre des mesures liberticides ! S'ils avaient été au pouvoir, la vaccination aurait perdu des mois et les morts auraient été bien plus nombreux, comme chez leurs amis Bolsonaro l'antivax ou Poutine, dont le vaccin inopérant était réclamé à grands cris par Mélenchon alors que même les Russes n'en veulent pas ! Les Français n'auraient eu droit Les Français n'auraient eu droit qu'aux remèdes bidons d'un gourou rocambolesque, validés par la Twitter School of Medicine et la Facebook University ! Ces stakhanovistes de l'erreur et du cynisme sont opposés au passe vaccinal, non pas pour préserver la santé de nos concitoyens, mais pour récupérer les voix des extrémistes. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux vous ferez mal ! Je vous suggère une idée : pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel, interdisez le vaccin, ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter Maintenant, cela suffit ! À 300 000 cas par jour, il est temps de répondre ; il est aussi plus que temps de faire front. La démocratie, ce n'est pas s'agenouiller devant une minorité inconsciente qui peuple aujourd'hui les services d'urgence et qui fait pleurer de rage et d'épuisement les soignants voyant leurs lits remplis de patients qui n'auraient jamais dû s'y trouver et qui en chassent tous les autres. La démocratie, ce n'est pas écouter des rebelles de supermarché sauter comme des cabris avec leurs pancartes en criant : « Liberté ! que j'ai passés comme médecin dans les guerres ou les épidémies, j'ai tiré une leçon simple : ce sont les virus qui bafouent les libertés et non les vaccins. Et si l'on ne prend pas les mesures qui s'imposent, c'est l'épidémie seule qui en décide, toujours de la façon la plus violente et la plus létale. létale. Comme il n'y a pas de liberté absolue, il faut trouver un équilibre entre des libertés contradictoires et prendre les bonnes décisions, même si elles ne plaisent pas à tous. C'est ce que vous proposez aujourd'hui, monsieur le ministre, et c'est ce que nous allons faire avec vous. Oui, le passe vaccinal est une façon de pousser à la vaccination. Pour tout dire, l'idéal serait la vaccination obligatoire : il en existe onze autres sans que personne ne hurle à la tyrannie monsieur le ministre, parce que vous craignez que les boutefeux ne finissent par déchirer un pays exténué et parce qu'en démocratie il n'y a pas de moyen infaillible de l'imposer ; vous avez sans doute raison. Alors, va pour le passe vaccinal ! Les offusqués professionnels diront que vous créez deux catégories de Français, alors que ce sont eux qui se placent en marge et nous mettent en danger. Ils diront que vous les stigmatisez, alors que depuis un an ils traitent les vaccinés de moutons et les soignants de collabos, alors qu'ils menacent de mort les élus et saccagent leurs permanences. Mais nous allons poursuivre ensemble, calmement, la lutte contre l'épidémie, malgré eux et avec l'immense majorité des Français ! Oui, car en dépit des campagnes incessantes sur les réseaux antisociaux, les Français ont montré une remarquable compréhension, une remarquable patience et une remarquable responsabilité. Malgré les intox, la France est dans le peloton de tête des pays les plus vaccinés. Les réseaux ont même eu une vertu : après deux ans de bobards, nos concitoyens ont fini, devant l'énormité des, par se faire une solide opinion sur ceux qui les diffusent et je préfère ne pas répéter ici les épithètes dont ils les gratifient. Quant aux discussions dans les repas de famille où se trouvait un antivax pendant les fêtes, elles ont définitivement vacciné des millions de Français contre les absurdités. Or ce vaccin-là, par chance, est d'une grande efficacité

Or nous voici, au début de 2022, encore en pleine pandémie : notre peuple fait face avec courage, mais aussi lassitude et résignation. il faut lutter frontalement contre l'épidémie ! Oui, il faut vacciner et protéger la population ! Mais deux ans après le début de l'épidémie, monsieur le ministre, vous ne pouvez plus dissimuler la réalité : c'est l'insuffisance des moyens alloués à la santé publique qui pousse à la mise en oeuvre de politiques autoritaires et de contraintes qui portent lourdement atteinte aux libertés publiques. C'est l'hôpital public, la médecine de ville mais aussi l'assurance maladie qui sont défaillants,

Vous masquez par des mesures coercitives, comme le passe sanitaire, puis le passe vaccinal, et par l'état d'urgence permanent, l'incurie d'un système qui a ravalé la santé au rang de marchandise. Je le souligne d'emblée si le passe sanitaire a boosté la vaccination, force est de constater qu'il n'a pas ralenti la propagation du virus. Bien sûr ! Pour preuve, 300 000 personnes sont testées positives chaque jour : quelle est donc l'utilité de ces sésames ? Ce rideau de fumée, c'est aussi l'agression verbale du Président de la République contre des millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, souvent non pas par choix, mais par éloignement, faiblesse ou incompréhension. Quelle est cette France où l'on sonde les gens pour savoir si les soins doivent toujours être accordés à ceux qui refusent le vaccin ? Vous fabriquez des parias pour détourner le débat. Nous dénonçons ce jeu dangereux

ce passe a pu être utile, faute de politique de santé publique efficace pour inciter à la vaccination, on peut aujourd'hui se demander ce qui légitime sa prolongation et son durcissement.

de mettre fin à ce système de passe, à la fois inutile du point de vue sanitaire et dangereux pour les libertés publiques. Bien d'autres solutions sont possibles, des solutions d'ordre véritablement sanitaire et non sécuritaire,

l'organisation de roulements dans les entreprises ou dans les établissements scolaires. Plus globalement, il conviendrait, comme nous n'avons de cesse de le réclamer, d'investir davantage dans la médecine de ville et la médecine scolaire et de réarmer l'hôpital public. En bref,

le problème est donc mondial et la seule réponse efficace sera à cette échelle. C'est pourquoi, je le redis, il est plus urgent que jamais de lever les brevets sur les vaccins si l'on veut éviter l'émergence de nouveaux variants.

du poing sur la table en insultant toute une partie de nos concitoyens, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à profiter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour convoquer un sommet international et engager un bras de fer salutaire autour de la levée des brevets sur les vaccins et d'un gigantesque effort d'aide au développement. En France, nous avons débloqué des centaines de milliards d'euros pour l'économie, mais combien pour la santé, combien pour la solidarité internationale ? Mes chers collègues, monsieur le ministre, vous en conviendrez, nous sommes prêts à être une force de proposition et à débattre des mesures de nature à gérer la crise sanitaire. Mais, pour l'heure, malgré les tentatives du rapporteur de la commission des lois lois d'atténuer certaines mesures, nous nous opposons à ce énième projet de loi sécuritaire, d'intimidation et d'infantilisation de nos concitoyens et de déresponsabilisation de nos dirigeants. Emmanuel Macron avait annoncé, le 12 mars 2020, extraire la santé de la loi du marché. Or il fait aujourd'hui payer à notre peuple au quotidien, par ses décisions solitaires, le refus de s'attaquer aux dogmes libéraux qui étouffent l'hôpital, la santé et notre pays. Nous refusons cette impasse sanitaire, mais aussi démocratique.

ce texte n'aura pas d'effet sur les vagues en cours, sur la désorganisation de la société, sur le drame d'une école maintenue ouverte coûte que coûte au lieu d'être sécurisée coûte que coûte. Ce texte ne répond pas à une nouvelle urgence sanitaire ; il n'est pas destiné à freiner la propagation du virus. Ce n'est pas son objet.

La droite sénatoriale roumègue, mais vote toujours en essayant d'encadrer périmètre et durée. Nous sommes donc en état d'urgence perpétuel : sécuritaire hier, sanitaire aujourd'hui. Quoi vous focalisez sur des objectifs dérivés : lutter contre le reconfinement plutôt que contre l'épidémie, sauver Noël plutôt que notre système hospitalier. Derrière vos « choix d'équilibre », il y a au mieux un attentisme optimiste, au pire un critiquable calcul politicien.

Cette vision séparatiste de la société, triée par les passes successifs, nous la rejetons. Nous y sommes totalement opposés. Ce passe vaccinal n'empêchera pas la transmission et la propagation du virus, faute de moyens contraints alternatifs, comme les tests PCR ou les masques FFP2.

comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer ici, son efficacité en tant que telle, c'est-à-dire son simple pouvoir de limiter l'accès des personnes non vaccinées à certains lieux de vie, est peu étudiée et encore moins quantifiée à moyen terme. C'est pourtant ce pouvoir qu'il faudrait juger aujourd'hui.

Qui plus est, une partie du public prioritaire n'est toujours pas bien vacciné. Les plus fragiles, les plus précaires, les plus pauvres, les plus éloignés de l'épicentre de notre vie sociale ne le sont pas suffisamment et ce ne sont pas des antivax. Le passe vaccinal aura-t-il un effet protecteur sur ces populations ?

serait de protéger davantage la population sans devoir recourir à des mesures de restriction généralisées, dans un contexte où la vaccination est le meilleur outil pour lutter durablement contre le virus. virus. Néanmoins, comme l'a souligné le rapporteur, ce texte n'est pas une réponse à l'urgence sanitaire ; ce n'est d'ailleurs pas son objet. Il ne va pas réduire le rythme de circulation du variant omicron à court terme. terme. Sa mesure phare, le passe vaccinal, qui se substituerait au passe sanitaire, n'est pas sans poser quelques questions à nombre de nos concitoyens.

Ceux qui sont radicalement opposés au vaccin seront-ils plus convaincus par le passe vaccinal qu'ils ne l'ont été par le passe sanitaire ? C'est la question qui se posera

face à cette accumulation de mesures prises par le Gouvernement et aux contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres, mesures qui viennent parfois se contredire d'une semaine à l'autre. Je pense tout particulièrement aux enseignants, aux parents d'élèves, aux dirigeants associatifs, aux acteurs du milieu culturel. Comme je peux les comprendre effet, monsieur le ministre, votre péché originel, c'est votre méthode de communication, qui peut parfois paraître totalement incongrue au regard des annonces faites.

de consommer du pop-corn au cinéma, de boire son café debout, ou encore sur l'annonce du retour des fameuses jauges pour les événements culturels ou sportifs, qui ne sont pas proportionnées à la taille des enceintes, j'ai envie de vous dire : tout ça pour ça Cela pourrait sembler anecdotique, si cela n'entravait pas la bonne gestion de la crise sanitaire en jetant notamment le doute sur l'efficacité de l'action publique et sur la nécessité de poursuivre l'effort vaccinal.

Je ne le pense pas : ce serait totalement irresponsable au regard de la situation sanitaire. Le Sénat a d'ailleurs toujours fait preuve de responsabilité et a toujours agi dans une logique constructive et rationnelle.

au Gouvernement, dès lors que la situation épidémique s'améliore, celle-ci étant mesurée par des critères cumulés- le niveau d'hospitalisations à l'échelon national, une circulation faible du virus et un taux de vaccination très élevé à l'échelon local. Cette disposition permettra ainsi de garantir une proportionnalité entre les limitations des libertés individuelles et la réponse à l'urgence sanitaire.

Troisièmement, concernant le renforcement des dispositifs de contrôle et de sanction, nous avons une conviction forte : ce n'est pas la vocation des restaurateurs, des hôteliers, des cafetiers, en somme de toute personne chargée des contrôles au sein des établissements recevant du public, de jouer le rôle d'officier de police judiciaire en contrôlant des cartes d'identité ou en identifiant des faux. La commission a donc strictement limité cette disposition, mais c'est un point qui, sans nul doute, fera débat au sein de notre hémicycle lors de la enfin, nous avons supprimé l'institution d'un régime de sanction administrative pour les entreprises ne respectant pas certaines préconisations sanitaires telles que le télétravail. Ce dispositif coercitif, qui laisse à l'inspection

la position d'équilibre et de cohérence qui a été la sienne durant la crise, afin de garantir la conciliation des objectifs de lutte contre l'épidémie, de préservation des libertés publiques et d'efficience du contrôle

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Parlement n'est pas le greffier de l'exécutif.

fait des innombrables mails que vous avez peut-être reçus les uns et les autres. Je vous propose de relativiser : le passe vaccinal est un passe sanitaire

? Voilà qui explique que vous soyez saisis pour la douzième fois, mes chers collègues ; M. le ministre et l'orateur précédent l'ont souligné. C'est finalement l'idée que le Gouvernement doit prouver qu'il agit et protège

Pour le groupe Union Centriste, la priorité est la santé publique. La pression du covid-19 est considérable, chacun peut la mesurer autour de lui, au-delà des statistiques qui ont été rappelées. Au-delà des personnes atteintes, vous avez pu mesurer la réalité des covid longs ou la réalité des formes dures que telle ou telle de vos relations a pu subir sans être forcément hospitalisée : le virus est en effet très lourd et très dur dans ses conséquences. Même avec un variant moins virulent, le risque pour nos concitoyens et pour le système hospitalier est majeur. La réponse est connue de tous : c'est la vaccination.

C'est ce qui explique que, très majoritairement, avec la liberté de vote qui lui est traditionnelle, notre groupe approuvera le passe vaccinal,

C'est dire si la clause de caducité est fondamentale. Le passe sanitaire doit être et rester exceptionnel, il doit avoir une fin. Le rapporteur a avancé une proposition combinant nombre de patients hospitalisés, taux de vaccination et taux de circulation Sous réserve d'ajustements sur ces critères ou sur la durée, notre groupe est très favorable à une clause de caducité ou d'extinction automatique du passe sanitaire et non à la seule référence à la date du 31 juillet

a été dure avec la jeunesse de France depuis deux ans. Nous partageons l'objectif de la commission des lois de donner plus de souplesse

nous sommes ouverts à la discussion. Le rapporteur a proposé qu'il n'y ait pas de vérification de la carte d'identité et qu'il soit possible de présenter d'autres documents portant une photographie nous ne voyons pas très bien à quoi correspondrait cette situation et, plus généralement, nous pensons qu'il y aura très peu de situations dans lesquelles, par exemple, un restaurateur estimera qu'il y a une raison sérieuse d'aller au-delà de la production du passe sanitaire. En résumé, nous restons ouverts à la discussion,

au risque de provoquer un arrêt de son activité. Nous ne voyons pas de raison de renoncer à cette situation de confiance et d'entrer dans une logique de sanction. Reste pour moi à évoquer un autre sujet,

vous le savez tous, l'élection présidentielle est la clé de voûte de nos institutions. Alors que des dispositions ont été adoptées pour faciliter le vote aux élections

et élargir la campagne à la télévision. Nous la soumettrons à tous les groupes de cette assemblée, mais nous souhaitons auparavant connaître la position du Gouvernement sur cette question. Je terminerai en évitant d'ajouter ma petite phrase à toutes celles qui ont déjà été prononcées sur les déclarations des plus hauts responsables

après les tumultes que ce texte a pu susciter la semaine dernière- que les perturbations viennent de l'exécutif ou de parlementaires -, le Sénat peut enfin se pencher sur la question du passe vaccinal.

Nous voyons dans nos départements combien les hôpitaux sont débordés et leurs personnels épuisés. Nous sommes également peinés de voir des familles endeuillées, alors que certains patients, s'ils avaient été vaccinés, auraient pu guérir de cette maladie. Oui ! Nous connaissons de mieux en mieux le virus, son mode de fonctionnement et ses effets.

Il faut donc trouver le moyen le plus opérant pour achever cette campagne vaccinale. Faut-il durcir l'incitation, comme le propose le Gouvernement au travers du nouveau passe ? Faut-il penser un nouveau mécanisme d'obligation, comme le suggèrent certains ? Bien entendu, le texte idéal n'existe pas et chacun trouvera toujours à redire sur le dispositif choisi. Ce qu'il faut éviter, c'est l'immobilisme. Certains membres du groupe du RDSE se sont très tôt prononcés en faveur de l'obligation vaccinale au point qu'aujourd'hui, avec ce nouveau passe, nous nous interrogeons sur l'intérêt de maintenir un faux-semblant de liberté de choix. Il est sans doute trop tard, mais un autre dispositif aurait pu être imaginé en amont, par exemple afin d'épargner aux restaurateurs et aux cafetiers toutes ces contraintes quotidiennes, que nous pourrions d'ailleurs encore alourdir en leur ouvrant la possibilité de vérifier l'identité des détenteurs de passe. Il demeure que le chemin du passe sanitaire a été choisi et que nous poursuivons dans cette voie. Reste à espérer que ce mécanisme permettra de convaincre ceux qui, pour des raisons qui leur sont propres, refusent encore d'être vaccinés. Nous devons néanmoins garder à l'esprit la nécessaire mesure que ce type de dispositif requiert. Après quelques mois d'utilisation du passe sanitaire, nous nous sommes accoutumés. Cela suscite une première inquiétude : cette banalisation pourrait conduire à un usage excessif. je ne vous apprendrai rien en rappelant qu'une mesure administrative intervenant en matière de police générale n'est légale que si l'atteinte portée au libre exercice des droits et libertés de chacun est adaptée, nécessaire et proportionnée. Ce principe s'impose à l'administration, donc au Gouvernement, mais il doit aussi guider le législateur lorsqu'il fixe le cadre de l'exercice de cette police administrative, en lui imposant de respecter une proportion équilibrée entre la gravité de l'atteinte portée aux droits et libertés et l'intensité du risque encouru, en l'espèce sanitaire. C'est une exigence de l'État de droit. Aussi, nous devons tenir compte des situations spécifiques et ne pas céder à la facilité d'imposer des obligations trop générales, au seul motif qu'elles sont commodes à appliquer. Dans ces circonstances, le texte adopté par l'Assemblée nationale nous paraissait encore perfectible. Par exemple, la question de la proportionnalité des mesures se pose encore une fois, à l'heure où les jauges ont été rétablies dans de nombreux lieux culturels. L'Assemblée nationale a fait un pas vers plus de flexibilité lors de l'examen du texte en commission, nous regrettons qu'elle soit revenue sur son intention en séance publique.

Dans l'ensemble, les amendements adoptés en commission vont dans le sens que nous attendions : ils visent à assurer un meilleur encadrement juridique du passe vaccinal de sorte qu'il ne donne pas le sentiment d'être un outil auquel tout gouvernement pourrait recourir sans difficulté.

objectif de soigner, ni même de protéger les Français. Son objectif n'est plus sanitaire, il est politique. Il veut tout simplement donner l'illusion de faire quelque chose en prenant la décision la plus arbitraire et autoritaire que ce pays ait eu à subir depuis trois quarts de siècle. Si son objectif était de protéger nos compatriotes, il rendrait les tests gratuits pour tous, il investirait massivement depuis deux ans dans l'hôpital et la recherche. Or rien de tout cela n'a été ne serait-ce qu'amorcé. Tout vaccinés que vous êtes, mes chers collègues, je suis le seul le seul à m'être fait tester ce matin- et je suis négatif ! Je suis en mesure d'affirmer que je ne contaminerai personne ici. Qui, dans cet hémicycle, peut en dire autant ? La dérive autoritaire est terrifiante et ce qui me terrifie encore plus, c'est la docilité du Parlement- de l'Assemblée nationale hier et du Sénat aujourd'hui -, qui va avaliser vos décisions, monsieur le ministre, sans que presque personne y trouve à redire. à redire. Que les députés de La République En Marche soient des godillots, on le savait, mais que la majorité de droite du Sénat vote ce texte, sans prendre en compte les atteintes irréparables à nos libertés, c'est plus qu'inquiétant, c'est mortifère. Oui, vous êtes en train de martyriser la démocratie et la liberté. Vous faites de 5 millions de Français, dont je suis, des sous-citoyens, des non-citoyens. Qu'avons-nous fait pour mériter pareil châtiment ?

Nous n'en voulons pas ? Qu'importe ! Le ministre nous l'impose de façon déguisée, alors même que le Conseil d'État s'y est opposé en ces termes : Le passe sanitaire ne doit pas « être justifié [ ...] par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner ». C'est pourtant clair. Comme de l'État de droit vous vous moquez, vous devriez aller encore plus loin : il faudrait écarter les non-vaccinés du reste de la société, les éloigner des vaccinés, comme je l'ai été sur le plateau de LCI, La Chaîne Indigne.

Sachons nous rappeler la citation de Benjamin Franklin, qui correspond parfaitement à ce que nous sommes en train de vivre : « Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. » Mes chers collègues, en votant ce texte infâme, vous assassinez nos libertés sans assurer notre sécurité. Ce texte est une honte pour vous, pour la République et surtout- surtout ! -pour la France.

notre position a été claire : au mois de novembre dernier, à l'instigation de notre collègue Bernard Jomier, que je tiens à saluer, notre groupe a à l'unanimité l'obligation vaccinale. Parce que nous croyons en la science, parce que nous sommes le pays de Pasteur parce que onze vaccins sont déjà obligatoires dans notre pays, nous avons fait ce choix, en toute responsabilité. Nous le revendiquons et nous le maintenons. Nous étions le seul groupe à soutenir une

Si l'on avait opté pour la vaccination obligatoire des plus de cinquante ans au lieu du passe sanitaire en septembre 2021, on aurait évité 45 % des entrées en réanimation entre octobre et décembre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, 90 % des Français éligibles sont vaccinés, même partiellement je tiens à le souligner, car voilà un an, personne n'aurait osé espérer un tel succès. Le choix de la science, le choix de la responsabilité est toujours le bon. C'est celui qui a été fait par la grande majorité des Français. Certes, la vaccination n'empêche pas totalement d'être contaminé ou de transmettre le virus, mais elle réduit considérablement le risque d'être hospitalisé ou admis en réanimation, et même de mourir du covid. Un tel bilan est déjà très positif, même si la vaccination ne nous a pas encore permis de reprendre une vie normale. Nous considérons que celle-ci constitue l'un des meilleurs outils pour lutter contre les dangers de l'épidémie. Actuellement, le problème majeur est celui des effectifs à l'hôpital et de l'épuisement des soignants. La vague omicron n'en finit pas de monter. Le taux de positivité des tests a atteint un niveau inédit, 20 %. Toutes les régions et toutes les tranches d'âge sont touchées. La pression

Comment allez-vous faire face au manque de personnels au moment où le nombre d'hospitalisations progresse ? Les conséquences sont déjà lourdes pour les autres patients. Les déprogrammations pourraient être évitées si les lits de réanimation n'étaient pas occupés par des personnes non vaccinées. telle situation pose la question de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective en matière de vaccination. Face à un virus qui évolue constamment, il est nécessaire d'adapter les outils pour le combattre, mais il faut aussi anticiper. égard, monsieur le ministre, nous regrettons le manque d'anticipation de la part du Gouvernement. En effet, les personnes actuellement en réanimation sont majoritairement touchées par le variant delta, qui n'est pas apparu ces jours-ci. Le texte

Les services hospitaliers sont saturés, car 5 millions de Français ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Il nous faut poursuivre nos efforts en transformant le passe sanitaire en passe vaccinal et en renforçant les mesures de lutte contre la fraude. Nous proposerons aussi un certain nombre de mesures pour améliorer la protection de tous les Français face à l'épidémie. J'ai notamment proposé des amendements visant à maintenir et à renforcer la surveillance épidémiologique des eaux usées et à favoriser l'installation de purificateurs d'air dans les établissements d'enseignement. Malheureusement, ils ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. Le Gouvernement a fait le choix de laisser le virus circuler en ne repoussant pas la rentrée. Mais, avec le nouveau protocole et la multiplication des tests, ni les parents, ni les enfants, ni les enseignants ne savent comment faire.

Enfin, au lieu d'invectiver les non-vaccinés, quelles mesures proposez-vous pour aller vers les plus vulnérables, les plus âgés, les plus isolés et les plus précaires ? Nous attendons beaucoup des débats qui vont suivre pour améliorer la gestion de la crise sanitaire.

Et pourtant, le Gouvernement a tenté de passer en force, jusqu'à s'offusquer que les députés ne veuillent pas délibérer à quatre heures du matin. Très juste ! Il est compliqué- pourtant, pourtant, vous savez que nous ne sommes pas irresponsables en matière de gestion de la crise sanitaire -d'approuver un texte qui relève à ce point de la posture politique.

ne partagent pas l'opinion majoritaire et ne voteront pas le passe vaccinal. Beaucoup de choses ont été dites. Mais beaucoup de choses resteraient à dire, par exemple sur la manière dont ont été caricaturés ceux qui étaient opposés à la position du Gouvernement, avec des propos tenant parfois plus des pires travers des réseaux sociaux que d'une méthode digne de gouvernement. Très bien ! Beaucoup de choses resteraient à dire aussi

Beaucoup de choses resteraient également à dire sur l'étrange philosophie de société qui nous pousse à faire courir tous les risques d'un vaccin somme toute assez récent à nos enfants au lieu de convaincre les plus âgés de se faire vacciner.

le vaccin n'est que peu efficace. En tout cas, il ne permet pas d'atteindre l'immunité collective. Plus nous sommes vaccinés, plus nous sommes contaminés ; c'est une évidence sur laquelle personne ne revient. En revanche, et ce n'est pas un petit apport, le vaccin permet de limiter les formes graves de ce virus. Or, au bout

qu'il attaque frontalement l'État de droit. L'État de droit, c'est la fin de l'arbitraire. Or, aujourd'hui, on nous propose de punir des personnes parce qu'elles ne se vaccinent pas alors même qu'il n'y a aucune obligation vaccinale ; c'est tout à fait arbitraire ! Quelles que soient les envies de nos dirigeants, nous ne pouvons nous ne pouvons pas y être soumis. Voilà pourquoi, mes chers collègues, un certain nombre d'entre nous et un certain nombre de Français sont opposés au passe vaccinal.

Qui aurait pu prédire qu'un jour, nous aurions 350 000 contaminations en vingt-quatre heures ? Le seuil, surtout fixé dans la loi, est rigide et nous empêche d'agir. Toutefois, les dispositions actuelles relatives à l'application du passe vaccinal

». En octobre dernier, c'est bien de fous que l'on nous qualifiait lorsque nous proposions la vaccination obligatoire pour tous. Force est de constater, aujourd'hui, que les événements nous donnent raison. Nous avions raison bien avant vous, monsieur le ministre, vous qui étiez défavorable à notre proposition de loi. projet de loi arrive bien trop tard. Si vous nous aviez écoutés à l'automne dernier, nous n'en serions pas là. La cacophonie que ce texte a provoquée à l'Assemblée nationale est symptomatique du désordre ambiant.

Monsieur le ministre, si le Président de la République n'avait pas fait preuve de toute la verticalité qui lui sied depuis le début de son mandat, il aurait pu constater que notre proposition n'avait pour but que de protéger nos concitoyens. Nous voilà donc aujourd'hui réduits à débattre d'un texte qui semble n'être que l'antichambre d'une obligation vaccinale déguisée,

plus de la moitié de nos concitoyens sont prêts à supprimer le financement des hospitalisations des personnes non vaccinées. C'est une atteinte extraordinaire à notre

Vous leur faites porter, d'ailleurs, la responsabilité des problèmes de l'hôpital. Le Président de la République nous explique qu'il a préféré l'incitation à l'obligation. J'ignorais que, pour convaincre,

Laurence Rossignol a rappelé que le contrôle et la sanction sont de véritables questions, mais que celles-ci sont directement liées au principe. Avec le passe vaccinal sans obligation, vous inventez le contrôle sans le principe,

mais vous êtes contraint par la voie qui a été choisie depuis des mois. Pour ma part, j'appelle chacun à se prononcer en conscience et j'invite la majorité sénatoriale à

En tout état de cause, le passe vaccinal que vous nous proposez ne va rien apporter de nouveau aux 80 % de nos concitoyens ayant un schéma vaccinal complet- pour eux, Malheureusement, un certain nombre d'entre eux contractent tout de même ce variant, même s'ils ne développent que des formes légères de la maladie. Mais vous avez choisi de contraindre les 20 % restants.

Demilly, sur l'article. L'article 1 que nous nous apprêtons à examiner a donné lieu à des débats houleux à l'Assemblée nationale, parfois sans lien direct d'ailleurs avec l'objet du texte étudié- comment pouvait-il en être autrement dans un pays qui compte 66 millions d'infectiologues ? Pardon pour cette ironie qui contraste avec la gravité de la situation ... L'ampleur de la vague épidémique se confirme jour après jour, nos hôpitaux sont saturés, nos soignants sont épuisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je viens de voter l'amendement n° Et puis, il y a les faits et ils sont têtus. Ils me rappellent mes cours de mathématiques et la loi de Pareto, également appelée loi des 20-80. Les non-vaccinés représentent 20 % de la population, mais peuvent représenter jusqu'à 80 % des patients en réanimation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas non plus Vilfredo Pareto, qui est mort il y a cent ans, c'est la Société française d'anesthésie et de réanimation. Mes chers collègues, il y a justement cent ans, au laboratoire Pasteur a été découvert le vaccin bilié de Calmette et Guérin, le fameux BCG, qui a permis de faire chuter la mortalité due à la tuberculose. le rappelle, car, dans notre pays, onze vaccins sont actuellement obligatoires. Sans ces recherches et sans les obligations de prévention, la rougeole, la coqueluche ou encore l'hépatite B ferait encore des ravages dans notre pays. Depuis quelques semaines, j'ai le sentiment que nous sommes engagés dans un débat surréaliste. L'Institut Pasteur, dans une étude portant sur un an, estime que la vaccination réduit la transmission du virus de 40 %. 40 %. Ce taux s'approche de ceux du Conseil scientifique, qui a démontré que la vaccination réduisait le risque d'hospitalisation de 95 %, le risque d'infection de 60 % et le risque de transmission de 50 %. S'il y a bien des moments où l'union nationale pourrait ou devrait faire sens, c'est bien face à des drames comme celui que nous traversons. Celui qui vous parle a passé un long séjour en réanimation, pour tout à fait autre chose. Je ne souhaite à personne de connaître les conséquences physiques, cognitives et psychologiques d'une telle déconnexion. Parce que je suis effectivement nourri d'une douloureuse expérience personnelle, parce que je suis outré de l'attitude de ceux qui oublient que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, parce que je considère que rejeter ce texte serait une insulte à la communauté scientifique, je voterai l'article 1 et l'ensemble du projet

nous avons aujourd'hui suffisamment de recul pour constater que ce seul outil n'est pas assez efficace, alors même que 90 % de la population éligible est vaccinée. Vous conviendrez avec moi, je l'espère, que les résultats promis et attendus ne sont pas atteints, notamment en termes de durée, et que la troisième dose ne mettra pas fin à la circulation du virus. Et pourtant ! C'est exclusivement sur cet outil que reposeraient demain la santé et la vie des Français. Jusqu'à l'absurde, puisque les gens vaccinés, mais testés positifs, pourront accéder à tous les lieux de contamination, tandis que les non-vaccinés testés négatifs devront, Précisons que ceux que vous appelez désormais les « non-vaccinés » comprennent les vaccinés ayant reçu deux doses. J'ai une pensée pour ceux qui ont subi des effets secondaires graves et que l'on traite aujourd'hui de « non-vaccinés », puisque c'est devenu une insulte, y compris dans la bouche du Président Il n'y a pas de citoyens irresponsables et encore moins de non-citoyens dans cette crise sanitaire. En revanche, il y a une stratégie du tout vaccinal qui ne fonctionne pas. Car, si c'était la faute des non-vaccinés, ce phénomène de fortes contaminations devrait être logiquement encore plus virulent dans les pays voisins, moins vaccinés que nous. Or ce n'est pas du tout le cas, ce qui démontre à la fois l'échec du passe sanitaire et l'inutilité d'instaurer un passe vaccinal. Non seulement je doute que ce projet de loi ait un réel intérêt sanitaire, mais je crains surtout ses effets délétères sur notre cohésion nationale et sur la vie de nos concitoyens, dont la santé ne se résume pas à avoir le covid ou non- j'y reviendrai lors de la discussion des amendements. La parole

atteindre un équilibre entre les mesures pour lutter contre le virus et la préservation de nos libertés. Cet équilibre, déjà fragilisé par le précédent projet de loi relatif à la crise sanitaire, est rompu par ce texte, qui- heureusement ! -a été revu, à bon escient, par les commissions. Pour lutter contre la covid, il est nécessaire de disposer d'une stratégie cohérente et rationnelle afin de proposer des mesures proportionnées et conciliables avec nos libertés. Or il semblerait que cette stratégie ne s'articule désormais qu'autour du souhait d'Emmanuel Macron d'« emmerder » tous les non-vaccinés, et cela au détriment d'une gestion équilibrée de la crise et de nos libertés. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'éléments suffisants pour établir avec certitude la pertinence de la mise en place du passe vaccinal.

La Défenseure des droits alerte sur l'absolue nécessité du caractère proportionné des restrictions. Or cet article 1 et l'obligation vaccinale déguisée qu'il cache ne répondent pas à cette exigence de proportionnalité. La vaccination, je suis pour, mille fois pour, bien entendu, mais pas à n'importe quel prix ! Nous disposons d'autres outils qui, utilisés judicieusement, permettraient de préserver nos libertés, tout en combattant l'épidémie. La

et qui n'ont pas pu rejoindre, par exemple, un parent mourant ou des proches en grande difficulté. Puis, l'introduction du passe sanitaire au début des vacances a bloqué ceux qui n'étaient pas vaccinés, parce que les vaccins n'étaient pas disponibles dans leur pays de résidence, ou ceux qui avaient reçu un vaccin non reconnu par la France, même s'il était par ailleurs reconnu par Nouvelle étape, le passe vaccinal réduit encore la liberté de mouvement de ceux dont le parcours vaccinal n'est pas reconnu. Pourtant, suivant les pays, les parcours et les avis des scientifiques diffèrent. Ainsi, au Japon, le délai imposé après la deuxième dose est de huit mois

D'autres solutions sont possibles. Il suffit de regarder comment certains pays sont arrivés à plus de 90 % de vaccinés sans créer de clivages ni de tensions dans la société, sans instaurer un contrôle permanent et par tous. Il eut été plus courageux d'assumer le principe de la vaccination obligatoire- nous venons d'en débattre -plutôt que de bricoler

Mais là aussi, il faut préciser clairement que les certificats de rétablissement établis par des autorités de santé de pays situés hors de l'Union européenne sont également recevables.

Les élus, conscients des conséquences des mobilisations successives, ont également rencontré des représentants des chambres consulaires, des socioprofessionnels, des chefs d'entreprise, des jeunes, des transporteurs de passagers et de marchandises, des personnes en situation de handicap et tous les tous les maires ou leurs représentants. Les élus de la Guadeloupe ont aussi échangé avec le ministre des solidarités et de la santé, le ministre des outre-mer, le Premier ministre et le Président de la République. Ils ont, pour la plupart, participé aux réunions du comité de suivi présidé par le préfet. Compte tenu de la situation sanitaire, sociale, économique, environnementale et systémique, les élus de la Guadeloupe ont également contribué à l'élaboration d'un amendement, lequel a été présenté à l'Assemblée nationale par les députés Benin, Mathiasin, Vainqueur-Christophe

de peser des principes proportionnés en amont d'un contrôle- ici, le passe vaccinal. J'en suis vraiment convaincu ! Or, avec ce texte et un passe vaccinal sans obligation vaccinale, nous ne sommes pas dans un État de droit

J'étais contre le passe sanitaire sans obligation vaccinale. De même, je pourrais être contre le passe vaccinal sans obligation vaccinale, obligation que vous venez de refuser. Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous avez lu l'avis de la Défenseure des droits, qui parle d'un rétrécissement des libertés. Nous sommes à l'heure d'un basculement populiste avéré, qui verrait la morale remplacer le droit. Nous sommes à l'heure où notre pays a plus que tout besoin d'unité et d'apaisement. Je ne peux pas m'associer à un gouvernement qui tente de créer des clivages, d'« emmerder » une partie de nos concitoyens. Vous préférez la morale au droit, monsieur le ministre ; alors, je vous laisse avec cette pensée dérangeante d'Hannah Arendt : « Ceux qui optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier qu'ils ont choisi le mal

Pour autant, la question essentielle reste posée : pourquoi faut-il passer du passe sanitaire au passe vaccinal ? À titre personnel, je n'en vois pas la logique, au moment où la pandémie s'envole.

Certes, on nous dit que, grâce au vaccin, on diminue le risque pour les malades de développer des formes graves de la maladie, mais pense-t-on réellement, mes chers collègues, que c'est en instaurant un passeport vaccinal

La vague omicron est là, elle nous dépasse. La virulence de ce nouveau variant est telle que le Gouvernement, de toute évidence, hésite sur la conduite à tenir, comme en témoignent les atermoiements sur le protocole le ministre, dans le même temps, vous mobilisez le pays, le Parlement et l'opinion publique. Vous créez de vives tensions en pointant du doigt les non-vaccinés et en mettant en avant le passe vaccinal, alors que- chacun le reconnaît -cette nouvelle contrainte ne sera pas de nature de l'épidémie. Pourquoi cette obsession de batailler sur le passe vaccinal alors que tant de combats plus efficaces restent à mener pour résoudre cette crise sanitaire et pour endiguer l'épidémie ? En premier lieu, la levée des brevets

Des années d'un libéralisme encensé sans retenue ont désarmé notre société face à une menace que nous n'avons pas vue venir. Lits d'hôpitaux fermés, numérisation à l'excès de l'assurance maladie Cet article 1, même aménagé, établit un dispositif anachronique, en décalage avec la réalité, dont le seul objectif est de dévier le débat pour mieux contraindre- nous en sommes de plus en plus convaincus -et pour banaliser cette contrainte.

ce qu'ont fait les marins-pompiers de Marseille et les pompiers de Paris. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, ceux-ci ont été pleinement engagés pour faire face à la pandémie. Avec l'appui des élus locaux, ils ont cherché à développer des outils permettant de gérer et d'anticiper l'évolution de la situation épidémiologique. Dès l'été 2020, les marins-pompiers de Marseille ont commencé à mettre en oeuvre une technique d'analyse des eaux usées. Celle-ci, unique en Europe, sauf aux Pays-Bas, permet d'avoir environ une semaine d'avance sur la circulation active du virus. En effet, l'analyse régulière des eaux usées de Marseille fournit des éléments il est possible d'évaluer la situation de l'épidémie de covid dans notre ville. Le vice-amiral Patrick Augier, qui est à la tête des marins-pompiers de Marseille, indique que « la précision de ce dispositif permet de cibler en un temps record des zones de surveillance, et ainsi d'intensifier les moyens engagés par les acteurs de la crise, comme des évaluations sanitaires ou des dépistages, en fonction des besoins exprimés. Nous voyons dans les eaux usées à la fois des gens asymptomatiques et des gens malades. Nous voyons, par conséquent, tout le monde. Ce dispositif intervient en quelque sorte en amont pour compléter les autres données habituelles sur l'évolution du virus. Aussi, monsieur le ministre, au-delà du « quoi qu'il en coûte », nous vous demandons avec d'autres collègues issus de différentes travées, y compris du groupe socialiste,

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le passe sanitaire n'a pas montré son efficacité. Il suffit de constater les chiffres de contamination aujourd'hui. vous avez été incapable de justifier son efficacité et vous vous enfoncez dans un durcissement des mesures, qui relève désormais de l'absurde. Quand le Premier ministre annonce que les vaccinés contaminés pourront prendre le train, mais pas les non-vaccinés négatifs, dites-moi s'il est nécessaire d'être épidémiologiste pour comprendre l'absurdité de cette mesure ! Je ne voterai pas le passe vaccinal, non pas parce que je ne veux pas protéger les Français ou que je suis antivax- je suis médecin parce que je me refuse à pratiquer, comme vous, monsieur le ministre, la politique de la terre brûlée. Je suis un enfant du contrat social de Rousseau et je ne veux pas du contrat du crédit social que vous proposez. Par des manoeuvres dilatoires, le Président de la République a désigné un bouc émissaire. Or seuls ceux qui ne peuvent affronter l'échec en ont besoin ... La

La complexité de ces mesures, loin de permettre d'endiguer efficacement la pandémie, contribue à l'épuisement collectif de notre pays. Plus généralement, l'article 1 instaure une société de surveillance, exercée par une catégorie de citoyens sur une autre. restreint les droits des personnes non vaccinées et donne un sentiment de protection aux personnes vaccinées, qui conduit à l'abandon des gestes barrières dans les endroits confinés soumis au passe. Pour intensifier la vaccination, il faut convaincre et renforcer la politique de l'« aller vers ». Le taux de vaccination cache d'importantes disparités territoriales et la frilosité envers les vaccins à ARN messager est toujours très présente chez les personnes non vaccinées.

a déclaré : « On vaccine en ARN messager. Honnêtement, c'est le plus efficace, à date, dont on dispose. » Nous nous opposons à d'autres dispositions de cet article, comme le renforcement des modalités de contrôle du passe, le durcissement des sanctions et le prolongement de l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique jusqu'au 31 mars 2022. Enfin, nos institutions démocratiques sont éprouvées par la multiplication des états d'urgence. Le risque de pérennisation des mesures restrictives prises dans le cadre de ces régimes d'exception est avéré. Mes chers collègues, en ce qui me concerne, je voterai l'article 1. Nous devons, à mon sens, mettre en place un passe vaccinal, c'est-à-dire une obligation vaccinale quelque peu déguisée.

une nouvelle étape dans l'atteinte aux libertés fondamentales. Je ne prendrai qu'un exemple : le dispositif permet à de nombreuses personnes, restaurateurs, responsables d'établissement de loisirs, vigiles ou vigiles ou autres d'effectuer un contrôle d'identité, qui n'en est pas tout à fait un, bien évidemment, grâce aux artifices du Gouvernement, puis à ceux de la commission des lois, mais qui demeure dans les faits un contrôle. Aujourd'hui, la contrainte devient la règle. La prolongation et le renforcement du passe sanitaire sont symptomatiques de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où l'exception devient la norme et où, effectivement, les lois d'urgence entrent dans le quotidien

la vaccination et toutes les mesures qui peuvent aller dans ce sens, mais il faut inciter et rassurer les personnes qui sont encore inquiètes et qui refusent de se faire vacciner. Cela doit être une priorité dans la gestion de la crise sanitaire.

Merci n° 9 rectifié. Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire prévoit de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. Sur quelles bases durcir les mesures et faire peser sur une minorité de Français de nouvelles restrictions, alors que le passe sanitaire, mis en oeuvre depuis plusieurs mois, n'a pas fait la démonstration de son efficacité pour lutter contre la contamination ? 90 % de la population française est vaccinée et les variants successifs se jouent des passes que l'on veut bien instaurer. Par ailleurs, sans méconnaître les apports de la vaccination pour les personnes âgées et fragiles, les virologues ne considèrent-ils pas comme un non-sens la vaccination de masse ? Le virus a évolué vers omicron, variant très contagieux

Le passe vaccinal signe aussi la mort sociale d'une partie de la population, qui n'est pas délinquante, puisqu'elle respecte la loi et qu'elle ne transgresse aucune interdiction législative. La citoyenneté de chaque Français doit-elle être tributaire d'une injection prodiguée tous les trois à

collègue. Il n'y a donc pas lieu de discriminer les Français en instaurant un passe vaccinal. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à prévoir la suppression de l'article 1 du présent projet de loi.

de ces mesures, qui nous paraissent à la fois discriminantes et liberticides. Nous préférerions une autre politique pour endiguer l'épidémie, incluant une aide et un soutien pour le personnel soignant épuisé, une aide et un soutien psychologique pour les jeunes, un moratoire sur les fermetures de lits, une généralisation des capteurs de CO2, une gratuité de la mise à disposition des masques, en particulier FFP2, une gratuité des tests,

Il pose une question de principe fondamentale que nous devons considérer avant les aspects médicaux, sanitaires ou scientifiques. Reculer un peu plus sur la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est confirmer que, depuis dernier, nous avons mis le doigt dans un engrenage mortifère de délitement de la cohésion nationale. Le tout vaccinal est à bien des égards contestable à court et à moyen terme d'un point de vue sanitaire, mais les conséquences du passe vaccinal à long terme sont surtout délétères d'un point de vue juridique et symbolique. L'objectif de santé publique ne justifie pas de recourir au tout vaccinal. Reculer sur nos principes, c'est accepter un changement de civilisation. Nos droits régressent, nous passons d'une société de libertés à une société d'autorisations. Monsieur le ministre, puisque vous nous faites pour une fois l'honneur de votre présence, permettez-moi de m'adresser à vous ! Le fait que vous instrumentalisiez la cause du covid ne signifie en aucun cas que vous détenez, seul, les solutions permettant de régler la situation sanitaire. Par cet article, vous assumez ne plus vouloir lutter contre la propagation du « virus », que vous supprimez de la loi, mais contre l'épidémie elle-même. Dieu vous entende ! Les conséquences juridiques de la suppression de ce petit mot sont lourdes : elles changent la nature des pouvoirs octroyés au Gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire. Par ailleurs, l'article 1 permet aux professionnels qui contrôlent les passes vaccinaux de leurs clients, qu'ils soient cafetiers ou restaurateurs, d'effectuer un contrôle d'identité, sans quoi les sanctions à leur égard pourraient être alourdies. J'ai envie de crier au fou ! Cette mesure est totalement disproportionnée sachant, par exemple, que les policiers municipaux dans nos communes n'ont même pas la possibilité de contrôler l'identité

De nombreuses informations contradictoires circulent, si bien que nos compatriotes sont fondés à se poser actuellement des questions auxquelles ils ne trouvent pas toujours de réponse dans les décisions qui sont prises par le Gouvernement. D'un côté,

ceux du pic de contamination du printemps 2021, mais ils s'en approchent. Près de 4 000 personnes sont entrées en service de soins critiques. Nous avons connu des périodes où l'on recensait jusqu'à 6 600 personnes

devant le Parlement ou de mobiliser des instruments d'action que vous avez déjà à votre disposition dans le cadre de la loi sur l'urgence sanitaire. Il faut en effet le dire, les chiffres qui attestent la gravité de la maladie chez un grand nombre de nos compatriotes sont là,

les chiffres, c'est un peu comme les lampadaires pour les alcooliques, cela sert plus à soutenir qu'à éclairer

mais la réflexion se doit d'être plus approfondie. Ainsi, les personnes non vaccinées n'enfreignent aucune loi. Le refus de cette vaccination est un droit, la possibilité de se faire soigner l'est aussi.

Chacun est libre de ses actes et de ses choix et ne doit pas risquer de se voir privé de ses libertés les plus fondamentales quand ils sont réalisés dans un cadre légal. Mais jusqu'où va la liberté ? C'est la question éthique principale

avant la fin de la session parlementaire,

en voilà une toute trouvée L'état d'urgence sanitaire n'a pas vocation à devenir notre régime juridique permanent. Le laisser courir pendant sept mois encore, sans aucune possibilité de contrôle, c'est accorder un blanc-seing à l'actuel gouvernement, ainsi qu'à celui qui sera constitué après l'élection présidentielle et dont on ne connaît pas encore les intentions.

du tout contrôle. Je m'inquiète devant la paresse intellectuelle qui conduit certains à tout relativiser. Les digues de la séparation des pouvoirs sautent ; le Parlement ne peut se dessaisir de sa compétence en matière J'ai bien compris, au vu des votes successifs intervenus cet après-midi, que vous cachiez votre proximité idéologique avec le Gouvernement derrière des circonvolutions juridiques. Comment pouvez-vous accepter, monsieur le rapporteur de la majorité de droite, que nous continuions à vivre dans ce régime hybride d'état d'urgence pérennisé ? En laissant filer cet état d'urgence, vous acceptez d'endormir le Parlement dans un véhicule dont le pilote continue de rouler à tombeau ouvert, pilote élyséen dont la pensée peu complexe en 2016 le conduisait à refuser de déchoir de leur nationalité les auteurs d'actes terroristes au prétexte que l'on ne traite pas le mal en l'expulsant de la communauté nationale, mais qui vante aujourd'hui la déchéance de citoyenneté pour les non-vaccinés

au mois de janvier et non au mois de février, de l'adaptation de ce régime, sur l'initiative du Gouvernement lui-même, qui a bien dû, compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, se ranger aux arguments que nous avions avancés au mois de novembre, c'est-à-dire que l'on ne peut pas gérer cette crise sans le vote d'une loi

vaccinal en voie d'extinction en fixant dans la loi des critères liés à la gravité de l'épidémie. S'ils étaient

pour lui l'adaptation à la réalité de la situation sanitaire et ne laisse pas les mains libres au Gouvernement- c'est bien notre objectif, n'est-ce pas ? -de maintenir le passe vaccinal si les conditions

La Défense Arena, stade du Racing 92, 2 000 spectateurs pour 30 000 places. Cette enceinte est effectivement considérée comme une salle de spectacle. Dans le même temps, un stade de 5 000 places pourra faire le plein, tout comme une salle de spectacle de 2 000 personnes. Où est la cohérence dans cette décision ?

Le spectacle vivant et le monde sportif professionnel rencontrent, depuis près de deux ans, des difficultés financières très importantes, que les mécanismes de compensation n'ont pas suffi à endiguer.

dans certaines catégories d'établissements recevant du public, en fonction des capacités d'accueil de ces établissements, plutôt que de définir des jauges en valeur absolue, ce qui ne répond, en fait, à aucun critère objectif d'évitement de la propagation du virus. Cette mesure avait d'ailleurs été adoptée par la majorité présidentielle en commission à l'Assemblée nationale. Elle permettait d'objectiver et de proportionner les jauges, avant que le Gouvernement ne choisisse d'associer, à cette notion de capacité d'accueil, la situation sanitaire et l'ensemble des caractéristiques- non objectivables -de ces établissements.

C'est ce que nous avons essayé de faire au sein de la commission des lois. Nous avons établi que la réglementation pour l'accès aux salles de spectacles et aux stades est « adaptée à la situation sanitaire »- cela va de soi -et « prend en compte les caractéristiques des établissements concernés »- grands ou petits

également se révéler inapproprié au regard de la diversité des configurations des établissements recevant du public. Deux établissements ayant les mêmes capacités d'accueil peuvent présenter des risques sanitaires différents selon les phases épidémiques ou les caractéristiques des variants contre lesquels nous cherchons à lutter.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants est parvenue à l'adoption d'un texte commun. La parole est à Mme Victoire